Nous avons toujours dit que nous préférions les introduire en deuxième lecture, pour avoir de la visibilité et pouvoir les calibrer au plus juste. Je vous proposerai, ce soir ou demain, d'actualiser l'article liminaire sur la base des prévisions

En effet, la crise du covid-19 a entraîné une forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Selon les prévisions du Gouvernement, cette hausse devrait atteindre 8,7 % au niveau national pour la seule année 2020. Cela représente un poids considérable pour les départements. Il est donc indispensable que l'État compense intégralement cette hausse des dépenses des départements en 2021, alors que les finances de ces derniers sont déjà largement mises à mal par les conséquences du covid-19.

Or, un certain nombre de départements risquent de voir leurs finances affectées par l'effet ciseaux résultant d'une baisse importante de leurs recettes de CVAE et de DMTO et d'une forte augmentation des dépenses de RSA. Il est donc proposé le versement par l'État d'une compensation aux départements concernés.

En effet, si un dispositif d'avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux, ou DMTO, a été prévu au titre de l'année 2020, aucun filet de sécurité n'est à ce stade envisagé pour 2021. Or, un certain nombre de départements risquent de voir leurs finances affectées par l'effet ciseaux résultant d'une baisse importante de leurs recettes de CVAE et de DMTO et d'une forte augmentation des dépenses de RSA. Il est donc proposé le versement par l'État d'une compensation aux départements concernés.

rectifié , qui sont relatifs à la situation particulière des communes forestières. Enfin, je demande le retrait des autres amendements. À défaut, mon avis serait défavorable.

Sincèrement, c'est scandaleux

pour les collectivités locales, au regard de dispositifs qui ont tendance à dégrader l'autonomie financière des collectivités locales.

tenir compte de la suppression partielle des impôts de production, donner des capacités aux entreprises, enfin attirer l'attention du Gouvernement sur des secteurs d'activité qui ont davantage

pour explication de vote sur les amendements identiques

Comment ne pas entendre ou comprendre l'objet de l'amendement ? Néanmoins,

aussi importante soit-elle, sur un territoire, en l'occurrence le département des Alpes-Maritimes. Je rappelle que,

à mettre en place un mécanisme de garantie du produit de la TVA au bénéfice des départements. Peut-être n'étions-nous pas les seuls ? Ce mécanisme se serait déclenché dès lors que le montant de la TVA affecté en année aurait été inférieur à celui qui a été versé l'année précédente.

Cela étant, je souhaite en dire un mot et solliciter le Gouvernement sur un point. En dépit des mises en garde réitérées des départements sur l'hypothèse de la survenance d'une crise au moins comparable à celle de 2008 ou de l'ampleur de celle que nous vivons actuellement, le Gouvernement n'a pas souhaité, dans le cadre de la compensation attribuée aux départements pour la perte de leur foncier bâti prévue en loi de finances pour 2020, garantir l'affectation d'un produit de TVA au moins équivalent à celui qui perçu l'année précédente. Il a en revanche fait adopter discrètement un amendement à l'Assemblée nationale pour éviter ce qui a été appelé, maladroitement je pense, un « effet d'aubaine » pour les départements.

nouvelle crise surviendrait. Nous souhaiterions savoir comment le Gouvernement entend anticiper une éventuelle perte de recettes pour les départements. Nous estimons que la mise en place d'une garantie pour préserver les finances des départements est nécessaire,

de se réduire en 2021. C'est donc un nouvel effet de ciseaux qui les frappe, tout comme les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, auxquels, d'ailleurs, on demande de participer à la relance par la commande publique, au moment même où leurs recettes- je pense à la CVAE, mais on pourrait aussi parler du versement mobilité -se dégradent ou sont incomplètement compensées. Lorsque le débat sur la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales a eu lieu ici, au Sénat, nous avons alerté le Gouvernement sur la nécessité de tenir compte du caractère cyclique des recettes de TVA.

sans accroître leur déficit. Enfin, l'adoption de cet article impliquerait finalement de contemporanéiser les versements de TVA aux collectivités locales, ce qui pourrait constituer un facteur important de fragilité, alors même que les garanties prévues sont particulièrement faibles. En conséquence, nous proposons

Le Gouvernement profite de la baisse de la TVA au titre de 2020, en raison de la crise sanitaire, pour caler le mécanisme d'évolution de la compensation sur la TVA au titre de 2021, aux dépens des collectivités.

proposons la suppression si l'on considère les choses très factuellement, en faisant complètement abstraction de la situation des départements, il y a bien un effet d'aubaine, la TVA de 2020 étant contractée.

Nous attendons des réponses concrètes, monsieur le ministre, puisque cet effet de bord positif pour les départements pourrait leur apporter 1 milliard d'euros, soit à peu près l'augmentation du RSA due à la crise

entraîne une réduction annuelle de la dynamique de compensation de l'État, à hauteur de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour les EPCI à fiscalité propre.

que les départements soient compensés par une fraction de TVA égale au montant de TFPB perçu en 2020, c'est-à-dire 15 milliards d'euros, et que les intercommunalités soient compensées par une fraction de TVA égale à

En 2022, d'après la loi de finances pour 2020, les départements devraient toucher 15,25 milliards d'euros, actualisés à hauteur de l'évolution de la TVA entre 2020 et 2021.

vise à tirer les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur les modalités de calcul et de répartition entre les contribuables de la taxe Gemapi, de la taxe spéciale d'équipement, la TSE, ainsi que des contributions fiscalisées des syndicats, comme le souhaite l'Association En effet, ces impositions sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux.

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a donc mécaniquement des conséquences sur ces dernières. Pour 2020, le taux additionnel issu de la répartition de la TSE, de la taxe Gemapi et des contributions fiscalisées sur la taxe d'habitation ne peut dépasser les taux appliqués en 2019.

de la TFB, de la TFNB et de la CFE. Cela a conduit, dans de nombreux cas, à une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables des taxes foncières et de la CFE, sur laquelle s'est reportée la part auparavant appliquée sur la taxe d'habitation, et ce même à besoins financiers constants. Ainsi, cet amendement tend à créer un prélèvement sur recettes de l'État, afin d'assurer une compensation de la fraction qui aurait dû être supportée sur la taxe d'habitation et de ne pas faire supporter sur une petite fraction des contribuables la totalité de la contribution à ces taxes.

qui n'ont pas été prises en compte par le Gouvernement et qui pèsent évidemment sur les communes et sur les élus locaux. Les impositions que sont la taxe Gemapi, la taxe spéciale d'équipement et les contributions fiscalisées des syndicats sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés par les conseils municipaux et communautaires. La suppression de la taxe d'habitation a donc des conséquences mécaniques sur ces impositions, qui y étaient adossées. Pour 2020, le taux additionnel, issu de la répartition de ces impositions sur la taxe d'habitation, ne peut dépasser les taux appliqués en 2019. La fraction restante du produit a donc été répartie entre les redevables des taxes foncières, ce qui a pu créer une augmentation

140 communes de Seine-Maritime seraient concernées par un tel manque. Nous demandons donc, conjointement avec de nombreux maires, qu'une compensation de l'État soit prévue pour assurer cette fraction, auparavant supportée par la taxe d'habitation. Quel

ni équitable. Il n'est pas nécessaire, parce que les communes peuvent décider de neutraliser le ressaut d'imposition foncière en rebudgétisant la contribution. est inéquitable, parce qu'un tel dispositif conduirait à réduire le montant des seules contributions fiscalisées, et non celui des contributions budgétaires versées par les autres communes membres du syndicat. Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de ces deux amendements.

de la réforme de la suppression progressive de la taxe d'habitation. C'est la raison pour laquelle il nous paraît opportun de prendre en considération le dernier taux voté, celui de 2019, pour l'application de cette réforme.

ce qui ne me paraît pas justifié. On savait depuis 2017, en effet, que cette réforme allait advenir et qu'elle ne serait pas compensée sur la base du taux de 2020.

ces derniers ne subissent pas de hausse d'imposition, de nombreux établissements publics de coopération intercommunale ont mené des politiques fiscales communautaires visant à augmenter leur taux de fiscalité, en lien avec une baisse de la fiscalité des communes. Ces communautés de communes ont d'ailleurs souvent utilisé des attributions de compensation, afin de compenser les pertes de recettes de TH des communes dans le cadre de ces politiques de neutralisation. Cependant, compte tenu de la suppression de la TH et de sa compensation figée au niveau du taux voté en 2017, plusieurs intercommunalités se trouvent dans des situations financières fragiles.

sont là les suites et conséquences des restructurations intercommunales, qui se sont évidemment accompagnées de dispositifs d'intégration fiscale. Lors de l'examen du PLFR 4, monsieur le ministre, vous avez bien volontiers reconnu que la mise en oeuvre d'une reprise financière au détriment des communes et des EPCI qui avaient fait varier leur taux de taxe d'habitation dans le cadre de ces dispositifs d'intégration fiscale

Ce mécanisme pose problème, en particulier dans le cas d'EPCI issus de fusions et qui ont dû mettre en place des mécanismes de lissage des taxes qu'elles prélevaient. Ces fusions ont causé des diminutions de taux sur certaines parties du territoire de l'établissement et des augmentations sur d'autres, décidées afin d'aboutir à un produit fiscal constant pour la nouvelle communauté, et cela sans prélèvement supplémentaire sur l'ensemble du territoire. Dans ces conditions- c'est ce qui nous importe -, la pression fiscale sur les contribuables reste stable sur le territoire, et l'augmentation du taux communautaire ne correspond qu'à une substitution fiscale de la communauté aux communes. Il n'est donc pas justifié d'appliquer un ticket modérateur qui pénaliserait un tel lissage, car le mécanisme institué ne prend pas en compte cette redistribution entre communes et communauté. tel ajustement peut avoir de graves conséquences pour certains EPCI et n'est pas conforme à l'engagement initial du Gouvernement de garantir aux communes le même niveau de revenus

sur deux points : d'une part, il ne vise que les ensembles intercommunaux qui ont conclu un accord de gouvernance financière, ce qui me semble trop restrictif

la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % de foyers les plus aisés. Paraphrasant les propos tenus par le Président de la République lors de son interview du 14 juillet dernier,

pour explication de vote.

au travers de cet amendement, une solution à la compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour les syndicats intercommunaux à vocations multiples,

qui regroupe douze communes ayant opté pour la fiscalité additionnelle, afin de mutualiser un certain nombre de compétences qui étaient auparavant exercées par chaque commune membre- je pense, par exemple, aux crèches et aux centres de loisirs. Ce syndicat levait la taxe d'habitation pour faire face à ses dépenses. Cette dernière ayant été supprimée sans compensation de l'État, le montant de la fiscalité additionnelle de 2021, imputé à la seule taxe foncière, ce qui entraînerait une évolution lourde de la fiscalité locale, touchant en premier lieu

la parole qu'il a donnée, à savoir compenser à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation.

il ne s'agit pas seulement des Sivom, mais de l'ensemble des communes qui ont fiscalisé leur contribution au syndicat de communes membres. Lorsque la contribution versée au syndicat est recouvrée comme une taxe additionnelle à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, la suppression de la taxe d'habitation se trouve susceptible d'entraîner, je le répète, un ressaut un ressaut d'imposition au détriment des contribuables fonciers. Cet amendement vise à neutraliser les conséquences de cette réforme pour les contribuables concernés en créant, à partir de 2021, une dotation de l'État, au bénéfice des syndicats de communes, de communes, égale, chaque année, au produit recouvré en 2020 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Il vise, corrélativement, à minorer chaque année le montant des contributions à recouvrer sur le territoire des communes concernées

début 2021, nous réunirons, comme c'est normal dans ce cas-là, la commission d'évaluation des transferts de charges entre l'État et les collectivités concernées pour les routes nationales. C'est à ce moment, sur la base des trois derniers exercices,

pour explication de vote. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre explication : ce n'est qu'une avance pour compenser le fameux transfert du réseau routier national concédé

Cette somme pourrait recueillir l'agrément des collectivités dans le cadre d'un régime usuel de transfert. Néanmoins, nous le savons, les conditions idéales ne sont pas réunies étant donné l'état d'entretien et de maintenance du réseau routier. Plusieurs rapports indiquent d'ailleurs que, pour éviter un état catastrophique du réseau routier national non concédé, il faudrait que l'investissement annuel de l'État passe de 600 millions d'euros à 1 milliard d'euros, et non à 800 millions comme c'est prévu.

sur un montant de 30 millions d'euros annuels. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à donner une suite favorable à cette discussion ? Comment allez-vous opérer pour inscrire dans un PLFR le montant annuel de 22,2 millions d'euros et pour verser une soulte de 7,8 millions d'euros sur une période minimum de cinq ans, durée qui permettrait aux collectivités de mettre à niveau avance de bien vouloir m'apporter ces éléments de réponse, en me précisant un délai. Je vous rappelle que, lors de l'examen de la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, qui verra le jour le 1 janvier prochain, le Gouvernement s'était engagé à compenser intégralement le transfert du réseau routier national non concédé par une dotation annuelle définie à hauteur du réel, avec l'accord des collectivités concernées, à savoir la CEA et l'EMS. le confirme, monsieur le sénateur, la procédure veut que l'on attende les conclusions de la commission d'évaluation des transferts de charges. Les chiffres que vous citez d'une estimation annuelle d'environ 22 millions d'euros sont des hypothèses de travail.

Compte tenu de la gravité de la situation, nos forêts ne pourront pas être entretenues ni replantées comme il se doit pour que le cycle de l'échange entre l'oxygène et le gaz carbonique conduise à une

pour créer un fonds d'amorçage en faveur des communes et des EPCI. Autant je partage la préoccupation exprimée, autant je pense que l'outil proposé n'est pas le bon, puisqu'il s'agit de financer de l'investissement avec des recettes de fonctionnement.

les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, qui font suite à nos débats passionnés et passionnants. Le dispositif proposé représente néanmoins une baisse de 9 % à périmètre constant,

également partie des principaux prélèvements en la matière pour nos collectivités territoriales : 6,5 milliards d'euros, avec une progression de 546 millions d'euros,

où non seulement l'ensemble des communes contribue, mais où certaines d'entre elles qui sont éligibles aux dotations de péréquation autofinancent celles-ci partiellement, voire totalement.

avec la suppression de la minoration des variables d'ajustement, à hauteur d'un peu plus de 37 millions d'euros. Du fait du même amendement, sont également majorées la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle,

d'un peu plus de 1 milliard d'euros, soit une hausse de 2,4 % par rapport au montant voté par l'Assemblée nationale et de 2,6 % par rapport au texte déposé par le Gouvernement.

n° I-1076 rectifié. Le Gouvernement a annoncé que tous les territoires seraient dotés de contrats de relance et de développement écologique d'ici à la fin de l'année 2021. Encore faut-il que ces contrats bénéficient de lignes de financements dédiés Or les besoins en financement du bloc communal pour l'investissement dans les seuls secteurs des transports, de l'énergie et du bâtiment ont été estimés par le think-tank Institut de l'Économie pour le Climat à 1,7 milliard d'euros annuels supplémentaires d'ici à 2023. Cet amendement vise à instaurer une hausse de 1,7 milliard d'euros de la dotation de soutien à l'investissement local au profit des collectivités territoriales, afin de leur permettre de mener des projets en matière de rénovation thermique, de transition énergétique ou de développement des énergies renouvelables.

un fonds qui, dans son fonctionnement actuel, se révèle une des plus grandes injustices fiscales créées, organisées et maintenues par un État. En effet, depuis qu'il a été figé en 2012, ce fonds, censé garantir des ressources, institue la spoliation officielle et méthodique de certains territoires. On prend à des communes devenues pauvres ce qu'elles n'ont plus. C'est un « anti Robin des bois », en quelque sorte ! Ces prélèvements ou reversements sont désormais fixes, sans tenir aucunement compte de l'évolution économique des territoires, c'est-à-dire des cessations ou des créations d'activités. On a ainsi des communes qui n'ont plus

Ce fonds, créé en 2010 afin de compenser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, présente l'inconvénient d'être figé. Or, parmi les collectivités contributrices, certaines continuent d'être prélevées au titre du FNGIR, alors que les facteurs expliquant cette contribution ont disparu. Tel est le cas, par exemple, de territoires qui ont connu depuis dix ans une forte désindustrialisation. C'est aussi la situation dans laquelle se trouvent la commune de Fessenheim et la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cet article constitue une solution d'attente pour régler cette difficulté. Il tend à prévoir que l'État verse annuellement la dotation égale à un tiers de la contribution du FNGIR aux communes et aux EPCI

pour des collectivités qui, comme la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, doivent s'acquitter d'une très forte contribution au FNGIR. communes continue d'être prélevée de près de 3 millions d'euros au titre du FNGIR, alors que la centrale nucléaire de Fessenheim a cessé de fonctionner.

pourquoi je proposerai deux amendements visant à accroître la prise en charge du FNGIR par l'État.

En attendant cette refonte en profondeur, qui se révèle nécessaire, et pour éviter de déséquilibrer le fonds tout en créant des difficultés nouvelles pour des collectivités qui n'en rencontraient pas jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement visant à apporter une première réponse provisoire. Il s'agit de mettre en place un nouveau prélèvement sur les recettes de l'État à destination des communes contributrices au FNGIR, qui ont connu depuis 2012 une perte de base de cotisation foncière des entreprises, de CFE, supérieure à 70 %. Cette mesure va indéniablement dans le bon sens, mais le Gouvernement s'arrête au milieu du gué, en ne prenant pas en compte les pertes de CVAE. Le présent amendement vise donc à combler cet oubli en remplaçant « cotisation foncière des entreprises par « contribution économique territoriale », ce qui permet de prendre en compte la CFE et la CVAE. En outre, le montant accordé se limite à seulement un tiers du prélèvement

Cette prise en charge serait alors intégrale. Serait concernée, notamment, la communauté de communes pays Rhin-Brisach, qui, je tiens à le rappeler, est en proie à un enjeu majeur de reconversion et de soutien à l'économie de son territoire, à la suite de l'arrêt des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim. Les collectivités ne pourront pas pleinement assumer le rôle majeur qu'elles ont à jouer dans cette reconversion si les effets du FNGIR ne sont pas neutralisés.

Simplement, à circonstance exceptionnelle, réponse exceptionnelle : il faut que l'État compense à 100 % cette communauté de communes. La fermeture de Fessenheim est

donner quelques éléments d'appréciation sur les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 23 Le fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, est un prélèvement sur les recettes de l'État, aujourd'hui évalué à 6,5 milliards d'euros et versé au profit des collectivités dont l'objet est de compenser ces dernières d'une partie de la TVA dont elles s'acquittent, notamment sur les dépenses d'investissement. Vous le savez, il existe trois régimes de versement des attributions du FCTVA : le premier, qui entraîne un versement l'année même de la dépense, représente à peu près 15 % du FCTVA

Je pense notamment aux dépenses de, que nous avons récemment rendu éligibles : les achats de matériel et de logiciels ont été remplacés par le recours à des solutions d'hébergement mutualisé.

J'en viens aux amendements qui tendent à augmenter le taux de compensation forfaitaire du FCTVA. Une telle mesure consisterait à augmenter le taux de ce fonds, ce qui ne me semble pas conforme à sa destination, puisque son objectif est de compenser la TVA acquittée, et non de la faire fonctionner comme une subvention. Enfin, des amendements ont pour objet de réformer les régimes de versement des attributions du FCTVA. L'existence L'existence des trois régimes de versement ne se justifie plus aujourd'hui, me semble-t-il. En revanche, les versements plus rapprochés de la dépense constitueraient une bonne et véritable incitation à l'investissement local. vous avez proposé plusieurs options pour réformer ce calendrier de versement du FCTVA. J'indique immédiatement que les amendements identiques n I-19 rectifié, I-596 et I-962 rectifié auront ma préférence.

Par ailleurs, ces amendements visent, me semble-t-il, à solder l'ensemble des attributions restant à percevoir en 2021, ce qui constituerait un utile gain de trésorerie au profit des collectivités locales. locales. Telle est ma position globale sur ces amendements, qui ont tous le même objectif : favoriser la relance et soutenir l'investissement des collectivités territoriales.

Cela favorise une gestion optimale du cycle de vie des produits et participe ainsi à la préservation de nos ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle il faut l'encourager. Aux collectivités territoriales qui recourent à la location de biens utilisés dans leurs opérations d'investissement, permet d'économiser des deniers publics et de mettre fin aux problématiques de stockage. Tel est le cas, par exemple, pour les engins de chantier. Ainsi, pour inciter les collectivités à y recourir, le présent amendement prévoit le remboursement de la TVA au bénéfice des collectivités, au titre de ces dépenses qui sont actuellement considérées comme des dépenses de fonctionnement. Il s'agit donc d'un amendement vertueux ! Quel est

Le Gouvernement souhaite favoriser la location longue durée de véhicules moins polluants, mesure [ ...] permettant d'étaler le surcoût à l'achat dans le temps et de favoriser la consolidation à court terme d'un marché de l'occasion des véhicules à faibles émissions. Afin d'enclencher cette dynamique pour les collectivités, le Gouvernement étudie le recours au fonds de compensation de la

Ensuite, nous prévoyons d'augmenter le taux forfaitaire, qui est actuellement de 16,4 %, pour le porter à 20 %, afin d'augmenter le volume de dépenses pris en charge pour les collectivités.

Les collectivités ont l'ambition d'y participer, mais cette volonté reste fortement tributaire de la baisse des recettes constatée en 2020 et attendue pour 2021, donc de leur grande difficulté à établir des budgets dans un contexte incertain.

Ainsi, pour une collectivité, la majoration de 100 % du taux du FCTVA s'appliquerait sur la fraction des dépenses éligibles qui dépasse la plus basse des compensations au titre du FCTVA lors des trois dernières années. Cette mesure s'appliquerait pour 2021 et 2022. Au titre de ce plan de relance, nous considérons que le FCTVA constitue un mécanisme tout à fait pertinent pour servir de support au soutien à l'investissement. Dans ce contexte, ce doublement du taux ne bénéficierait qu'aux collectivités souhaitant et pouvant s'engager dans la relance, de sorte que le fléchage de la dépense pour l'État vers celle-ci soit certain.

pendant la crise de 2009, lorsque le Gouvernement avait décidé d'anticiper, pour les collectivités qui participaient au plan de relance, le remboursement de la TVA. Nous sommes de nouveau, monsieur le ministre, dans une période de crise.

Depuis le plan de relance mis en place pour faire face à la crise économique de 2008, la majorité des collectivités perçoivent le FCTVA une année après la dépense ; certaines

qui avait prévu d'accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, notre proposition ne pose aucune condition en termes de volume d'investissement. Par ailleurs, cette mesure permettrait de simplifier la gestion du FCTVA pour l'État, en ne laissant subsister que deux régimes.

2021. Les collectivités relevant actuellement du versement en passeraient en tandis que celles touchant aujourd'hui le fonds en en bénéficieraient l'année même de la dépense.

sur la même base.

Cela s'articule difficilement avec le principe de dévolution du patrimoine des universités. Le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en élargissant le champ d'application de cette procédure, pour permettre aux établissements publics publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine de confier la maîtrise d'ouvrage selon les modalités prévues par le code de l'éducation.

l'État doit avoir confié, par convention, la maîtrise d'ouvrage de ses opérations à la collectivité ou au groupement de collectivités ; l'apport financier de la collectivité ou de son groupement doit être égal au moins aux deux tiers du coût, toutes taxes comprises, de l'opération réalisée ; les biens concernés doivent, à leur achèvement, être remis en pleine propriété à l'État. l'État. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le code général des impôts pour étendre aux établissements publics de l'État ce dispositif dérogatoire. Seules les dépenses d'investissement réalisées sur des biens appartenant à une collectivité bénéficiaire du FCTVA ou destinés à enrichir son patrimoine sont susceptibles, par ailleurs, de donner lieu à attribution du fonds. Il nous semble que prévoir une dérogation générale à cette règle au profit des établissements publics d'État créerait un précédent dérogatoire supplémentaire pour un dispositif que l'on aimerait simplifier et serait contraire aux intérêts financiers de l'État. Par ailleurs, cela dénaturerait l'objectif du FCTVA, qui est le principal instrument de soutien de l'investissement local de la part de l'État, notamment en période cyclique ou contracyclique. En outre, l'importance de l'élargissement induirait un véritable risque pour les finances publiques. La réforme du FCTVA automatisé, qui doit entrer progressivement en vigueur